L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2018, adopté par l'Assemblée nationale (projet Tous les crédits afférents aux missions ayant été examinés, le Sénat va maintenant statuer, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, sur les articles qui portent récapitulation de ces crédits.

de manière à tenir compte des votes qui sont intervenus lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances. Je mets aux voix l'ensemble constitué

cours de français, spectacles, services, prestations pour les candidats étudiants devant se rendre à l'espace Campus France, opérations de mécénat, Dans de telles conditions, la charge budgétaire constituée par l'emploi d'agents de droit local, recrutés à durée indéterminée ne repose pas sur le projet

entre un établissement à autonomie financière et un opérateur de l'État. Certains opérateurs de l'État, qui ne sont pas des établissements à autonomie financière, disposent de ressources propres. Néanmoins,

chers collègues, l'ACPR joue un rôle très important dans le contrôle du système bancaire et assurantiel français. Elle est chargée par la Banque centrale européenne d'exercer un certain nombre de contrôles sur les banques de faible et moyenne dimensions et elle surveille l'ensemble du système bancaire.

Pour toutes ces raisons, je propose de ramener le plafond d'emplois de l'ACPR à son niveau initial, c'est-à-dire à 1

Mme Nathalie Delattre. Nous le savons, avec le vieillissement de notre société dû à l'effet conjugué du et de l'allongement de l'espérance de vie, de nombreux proches viennent en aide aux personnes âgées et doivent de plus en plus souvent subvenir à leurs besoins. Le modèle de la famille traditionnelle a quasiment disparu. Toutes les générations ne vivent pas sous le même toit, mais dans bien des cas une ou plusieurs personnes de la famille s'occupent au quotidien de leur proche ou le placent dans un établissement spécialisé. Le modèle est différent, mais ce problème se pose également pour les familles des personnes handicapées. Je vous propose donc que l'article 156 du code général des impôts définisse le revenu imposable et les sommes qui peuvent en être déduites sous certaines conditions. Aujourd'hui, parmi les aidants de personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap, seuls les obligés alimentaires- ascendants ou descendants directs -peuvent bénéficier de ce dispositif de déduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils consacrent une partie de leurs amendement tend à déduire du revenu imposable les sommes versées par tout proche aidant de ces personnes dépendantes, en vue de leur maintien à domicile ou de leur admission dans un hébergement collectif de qualité. L'objectif est de permettre à tous les aidants de bénéficier de ce dispositif fiscal, en plafonnant la part des charges susceptibles de faire l'objet d'une déduction d'impôt à 30 % des revenus du proche aidant.

Autoriser une mobilisation immédiate du crédit d'impôt auprès d'un établissement financier du secteur privé faciliterait l'accès aux services à la personne du plus grand nombre de Français, dont les foyers les plus modestes, accentuerait la lutte contre le travail non déclaré, et entraînerait une simplification des procédures fiscales, le tout accompagné d'un renforcement de la lutte antifraude. En favorisant le recours à la consommation de services à la personne, une telle mesure participe en outre de l'amélioration de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. du présent amendement permettrait, à coût constant pour l'État, de simplifier la consommation de services à la personne, tout en relançant la consommation, en répondant aux besoins de services à la personne de la part des ménages, libérés de la contingence de l'avance sur consommation, et en soulageant la mobilisation de trésorerie des ménages, ménages, ceux des ménages à revenus modestes. Par ailleurs, cet amendement tend à s'inscrire dans l'universalisation du crédit d'impôt, la mobilisation immédiate de la trésorerie résultant du crédit d'impôt concernant tous les foyers, qu'ils soient imposables ou non. Un organisme consolidateur se chargera de vérifier les informations et de consolider les dépenses mobilisées pour s'assurer du non-dépassement des plafonds de la part des ménages, qui pourront bénéficier de ce dispositif directement ou indirectement, c'est-à-dire dans le cadre de l'emploi direct de personnel ou ou par le recours à des entreprises ou associations prestataires de services à la personne. Enfin, il convient de souligner que ce dispositif est à coût constant pour l'État, puisqu'il permettra une mobilisation immédiate des crédits d'impôt par les établissements financiers, restitution des crédits d'impôt par l'État dans les délais habituels de la liquidation de l'impôt sur le revenu, donc sans requérir d'efforts financiers de la part de l'État, ni en termes de montant ni en termes de calendrier de paiement. Quel est l'avis de la commission ? Nous avions déjà

de l'emploi dans ce secteur, avec un risque de rupture d'égalité et d'avantage concurrentiel en faveur des organisations qui offrent des services à la personne. Troisièmement, le dispositif proposé nous paraît juridiquement incertain, car la créance n'est ni établie ni garantie. compte tenu du plafonnement de ces dépenses, mais aussi du plafonnement global des niches fiscales ainsi que des aides à déduire, le montant du crédit d'impôt est trop incertain au moment du paiement de la prestation. Par conséquent, cette proposition n'est adossée à aucun mécanisme de garantie qui nous paraisse suffisant.

patrimoine, dite « LCAP », a permis en 2016 la création des sites patrimoniaux remarquables, les SPR, intégrant dans ce nouveau dispositif l'ensemble des outils existant s'appliquant aux espaces protégés paysager, ou ZPPAUP. Plus de 800 SPR ont été créés depuis sur ces espaces. Certains fonctionnent avec succès, mais d'autres connaissent de grandes difficultés. Dans la droite ligne des propositions formulées pour améliorer le dispositif par notre ancien collègue Yves Dauge, dans son rapport sur les nouveaux espaces protégés, commandé par Manuel Valls et remis au Premier ministre Bernard Cazeneuve, notre série d'amendements vise à rééquilibrer l'arsenal fiscal existant,

Un réajustement de la fiscalité permettrait, d'une part, de sauver un patrimoine menacé, et, d'autre part, de freiner le déclin des petites et moyennes communes qui, faute de moyens, voient leurs habitants quitter les centres anciens vétustes et leurs commerces et services fermer. Ce premier amendement vise à généraliser la déclaration d'utilité publique préalablement à l'attribution de la réduction d'impôt accordée au titre de la restauration des immeubles à usage locatif dans les centres anciens protégés par un SPR, selon le dispositif « Malraux « Malraux ». La DUP n'est aujourd'hui requise que si l'immeuble concerné par les travaux n'est pas situé dans un périmètre couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou par un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. En généralisant cette obligation de DUP, le dispositif fiscal Malraux ne s'appliquerait que de manière très sélective, dans les zones en SPR où le marché est amplement suffisant pour porter l'effort de l'investissement privé, c'est-à-dire dans de nombreux quartiers de grandes villes. Dans de tels quartiers, la fiscalité Malraux ne subsisterait que pour traiter certains points « durs », une fois les critères fondant l'utilité publique vérifiés. Cette restriction d'accès à la réduction d'impôt « Malraux » répond à un objectif de justice financière et une volonté politique de péréquation elle permettrait effectivement, en outre, de financer le dispositif, que nous présenterons dans nos amendements suivants, en faveur des communes moins riches qui ont besoin de dispositifs fiscaux plus attractifs pour revitaliser leurs centres anciens.

Delattre. Dans un pays où la forêt couvre 30 % du territoire, faut-il rappeler l'importance de son rôle ? Un rôle d'intérêt général reconnu par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, et renforcé par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Élue d'une région où la sylviculture contribue au dynamisme local, je connais bien les atouts de la ressource forestière, mais aussi ses faiblesses. Sur le plan écologique, nous savons qu'elle constitue un formidable captateur de C02. Sur le plan économique, la forêt concentre aujourd'hui environ 425 000 emplois, mais elle pourrait en générer beaucoup plus lorsque l'on sait qu'elle n'est exploitée qu'à 55 % de son accroissement. Aussi, sans méconnaître la portée des politiques publiques mises en oeuvre actuellement, notamment au travers de la signature de contrats stratégiques ou l'élaboration de plans tels que le Programme national de la forêt et du bois, je pense que nous pouvons faire plus. C'est pourquoi je propose cet amendement qui vise à renforcer les moyens du Fonds stratégique de la forêt et du bois en ouvrant le mécénat au renouvellement de la forêt dans le cadre d'une gestion durable effective. Hier matin, lors des débats consacrés à la mission « Agriculture », nos collègues rapporteurs ont souligné la faiblesse des crédits consacrés à la politique forestière pour 2018. S'agissant en particulier du Fonds stratégique de la forêt et du bois, si l'on souhaite atteindre l'objectif d'une capacité de mobilisation de ressources équivalentes à 100 millions d'euros,

au profit d'organismes d'intérêt général concourant à la défense de l'environnement naturel ouvrent d'ores et déjà droit à la réduction d'impôt prévue aux articles 200 et 238 du code général des impôts, comme l'a rappelé à l'instant M. le rapporteur général. C'est le cas des activités en faveur du renouvellement des forêts, qui participent à la défense du développement naturel. Pour être éligibles à cette réduction d'impôt, les dons et versements doivent satisfaire à plusieurs conditions et notamment être effectués sans contrepartie ou avec une contrepartie manifestement disproportionnée, en faveur d'organismes non lucratifs, qui, eux-mêmes, sont gérés de manière désintéressée et qui ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de particuliers.

De surcroît, en application de l'article 200 A du code général des impôts, une réduction d'impôt sur le revenu est aussi accordée au titre des cotisations versées aux associations syndicales autorisées qui ont pour objet la réalisation de travaux de prévention pour la défense des forêts contre l'incendie sur certains terrains. Cette réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées, dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal, et est exclue du champ d'application du plafonnement global des niches fiscales. Enfin, le régime fiscal applicable aux dons et versements

quelques remarques sur l'article 39, c'est-à-dire sur les dispositifs incitatifs au développement de l'offre locative. Dans un premier temps, ces dispositifs attirent plus ou moins l'attention des investisseurs, selon les caractéristiques propres à chaque produit, serais-je tenté de dire. On mesure l'importance du « cadeau fiscal », sa durabilité, ses effets secondaires éventuels- taxation des plus-values de cession ultérieures, obligations et contreparties -et la capacité d'y construire ou non un patrimoine plus ou moins important. Dans le cas du dispositif Pinel-Duflot, observons d'entrée qu'il s'agit d'un produit de défiscalisation supplémentaire. Le rapport général de l'Assemblée nationale nous indique que nous avons dépensé, en 2016, quelque 1 857 millions d'euros en dépense fiscale cumulée, dont l'essentiel porte sur le dispositif le dispositif Scellier, qui semble toutefois être arrivé à maturité, puisque la dépense est fixée depuis plusieurs années autour de 380 millions d'euros pour le dispositif « Scellier ordinaire » et au double pour le « Scellier intermédiaire Pinel-Duflot, pour sa part, est appelé à croître et embellir, puisque la dépense actuelle, de 191 millions d'euros, devrait passer à 554 millions d'euros dès 2018, grâce à la commercialisation d'un nombre croissant de programmes labellisés. Notons cependant ici, mes chers collègues, que pendant ce temps la ligne de crédit du budget de la mission « Cohésion des territoires », consacrée à la construction neuve et à la réhabilitation de logements locatifs ne comporte pour 2018 qu'un peu plus de 55 millions d'euros, et que l'on attend 425 millions d'euros de fonds de concours pour la compléter. Pour une partie, c'est-à-dire pour 375 millions d'euros, ces fonds de concours procèdent de la mutualisation forcée du secteur HLM, c'est-à-dire que le secteur HLM finance son propre développement Rapprochons d'ailleurs les 55 millions d'euros de crédits budgétaires de l'État sur la ligne de l'écrêtement de la taxe sur les logements vacants, et nous pouvons tirer la conclusion qui s'impose. Dans les faits, en 2018, l'État n'apporte plus son concours direct au financement du logement locatif social comme du logement en général. Il se contente d'accorder des facilités fiscales plus ou moins réelles aux investisseurs ou aux entreprises du secteur, tout en rechignant- nous l'avons vu avec la discussion de l'article 52 -à financer les aides au logement destinées aux occupants. Que fait l'article 39 ? Eh bien, il nous invite à prolonger cette expansion des travers actuels de la politique du logement en épuisant les possibilités du dispositif Pinel, destiné à créer une offre de logements intermédiaires pour les couches moyennes, dans la guerre spéculative des parties du territoire les plus tendues du point de vue du marché, et à délaisser, de fait, une partie importante du territoire, désormais privée de quelques-uns des maillons de la chaîne du logement intermédiaire.

Outre ces situations les plus graves, ce sont plus de 12 millions de personnes qui sont touchées à des degrés divers par la crise du logement. Tout d'abord, parmi les 896 000 personnes privées de logement personnel, une enquête de l'INSEE compte 143 000 personnes sans domicile. Le recensement de la population dénombre en outre 85 000 personnes en habitations de fortune, tandis que 24 733 personnes vivaient à l'hôtel en 2013, par exemple. Parmi les personnes privées de logement personnel apparaissent enfin 643 000 personnes hébergées chez des tiers de manière très contrainte. Ensuite, les mal-logés se composent de 2,819 millions de personnes vivant dans des conditions de logement très difficiles. On peut ajouter à ces chiffres les 39 000 résidents de foyers de travailleurs migrants en attente de rénovation, dans des conditions de vétusté parfois dramatiques.

C'est en ces termes que le vingt-deuxième rapport de la Fondation Abbé Pierre, publié en début d'année, fait état de la situation critique du logement dans notre pays. Aussi, recentrer le dispositif Pinel sur les secteurs tendus, c'est en fait drainer l'épargne des couches moyennes vers les programmes les plus complexes et les plus coûteux. De plus, c'est ignorer que l'outil a été utilisé pour 13 % dans des opérations menées en zone géographique C et pour moins de 3 % en zone A1, la plus tendue. C'est la zone B1, avec plus de 60 % des programmes, qui attire le plus le produit. D'où les motivations de fond qui sous-tendent Face à cette situation, il est grand temps de procéder à la création d'un nouveau dispositif d'accession à la propriété ou d'investissement locatif, qui partirait de la demande plutôt que de l'offre. Quel est l'avis de la

Nous considérons que, dans un contexte de crise du logement, cet instrument a contribué à la relance de la construction de logements dans le secteur intermédiaire et à la production d'une offre locative nouvelle. Ces effets positifs sont d'ailleurs reconnus par les professionnels du secteur de la construction, comme le démontrent les chiffres publiés

ce dispositif sur les zones géographiques où la tension entre l'offre et la demande de logement est la plus forte, en réservant le bénéfice du Pinel aux seules acquisitions ou constructions de logements dans les zones A, A et B 1 du territoire.

afin d'éviter une rotation par trop rapide de la propriété. Si l'on observe la situation actuelle, on constate d'ailleurs que c'est là la solution préférée des investisseurs.

on totalise 5 569 investisseurs avec engagement de six ans pour une quotité de 1 239 millions d'euros environ.

pour une durée plus longue, avec la possibilité de stabiliser la situation des locataires. Selon nous, neuf ans, c'est un bon compromis entre une proposition satisfaisant aux attentes des investisseurs une affectation du loyer à la location sur une durée suffisamment raisonnable pour pallier les travers de la précarité d'un bail de location d'aujourd'hui. Mes chers collègues, nous vous invitons donc à adopter cet amendement. Quel est l'avis de la

s'agit de rendre éligibles au dispositif fiscal Pinel, prévu par l'article 199 du code général des impôts, pour les investissements locatifs dans le logement neuf dit « intermédiaire », les travaux sur les immeubles en site patrimonial remarquable, Dans les centres anciens couverts par un SPR, il est parfois important de pouvoir reconstruire, quand l'habitat est devenu vraiment vétuste et insalubre, tout en préservant l'unité du quartier ou de l'îlot concerné. Il serait improductif de figer l'espace quand il n'est plus adapté aux exigences modernes de confort, de sécurité et d'esthétique. La revitalisation des centres anciens dont nous parlons doit être placée sous le signe de la diversité, et l'effort doit être porté vers tous les types de construction. Il faut absolument élargir l'assiette du Pinel à ces centres anciens classés SPR et reconstruire sinon, les habitants de logements anciens, humides et sombres continueront de migrer vers les périphéries qui leur offrent des logements neufs, dans des quartiers équipés, tous uniformes, et ce au détriment de ces centres anciens qui poursuivront leur lente agonie.

ont une grande responsabilité en la matière. Ils ont un rôle considérable à jouer pour atteindre cet objectif. Mais la fiscalité doit également être incitative. Le Pinel constitue, dans de tels cas, un outil adapté à notre vision globale de rénovation des centres anciens classés en SPR. Il permettra la reconstruction d'immeubles non pas destinés à une population de « nantis », mais à l'usage locatif dit « intermédiaire ». Aussi, cet amendement tend à s'inscrire dans un projet global patrimonial et sociétal.

le Pinel peut participer à des opérations d'aménagement urbain beaucoup plus complexes. Ces opérations associent la réalisation de logements neufs, en locatif social comme en locatif intermédiaire ou libre, sociale ou non, logements anciens réhabilités. Ce qui est essentiel, c'est que la palette de l'offre soit la plus diverse possible sur l'ensemble des territoires. Polariser le Pinel sur les zones tendues, c'est capter l'épargne des couches moyennes pour la cantonner dans le circuit de l'investissement spéculatif.

Évidemment, il ne s'agit pas de tout bétonner. Mais la demande en logements est une réalité. Je vous propose donc de proroger le dispositif existant pour une durée de deux ans, le temps de prévoir la transition qu'il exige.

sélection soit validée par le comité régional de l'habitat. Ce qui fut dit fut fait un peu tardivement : les décrets d'application et les décisions des comités régionaux de l'habitat n'ont permis

Nous proposons en effet de ramener ce montant de 300 000 à 200 000 euros, ce qui a été souligné : il semble bien, une fois encore, que le plafond en vigueur se révèle trop important au regard de la pratique. Partons des données disponibles.

le montant d'investissement atteint 200 560 euros pour les opérations avec engagement de neuf ans outre-mer et 169 800 euros en métropole. Le plafonnement à 200 000 euros est donc conforme à la pratique. Il ne fait que corriger la dépense fiscale Pinel des investissements les plus importants, qui n'ont peut-être plus grand-chose à voir avec le logement dit « intermédiaire ». Nous avons également exprimé notre intention de majorer d'au moins trois ans la durée minimale des engagements de location. Dans ce cadre, il n'est pas interdit de penser que la taxation ultérieure des plus-values de cession rapportera un peu moins qu'attendu aujourd'hui ; mais cet engagement prolongé sécurisera le parcours des locataires et donnera, de fait, une forme d'utilité sociale au Pinel. Cette utilité sociale ferait de cette offre de logements à loyers situés 20 % en dessous du marché un segment des parcours résidentiels. Nous proposons également de réduire le niveau de la réduction d'impôt.

tel calibrage du dispositif Pinel, qu'il s'agisse de l'engagement, de l'allégement fiscal et de la contrepartie, permettra de renforcer la pertinence de cet outil et d'en faire l'instrument des politiques d'aménagement urbain d'un grand nombre de collectivités

2017. Les logements qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire avant cette date pourront bénéficier du dispositif, à condition

donnons un coup de rabot brutal dans tous les éléments de politique, soit nous donnons du sens ! Au Parlement, on fait des choses parce qu'il y a du sens, et on a un projet pour notre pays.

un aménagement équilibré du territoire. Cessons d'opposer par des vues de l'esprit la ruralité à l'urbain ! Mes chers collègues, moi je ne comprends rien.

prochaine. Mes chers amis, nous n'arrêtons pas de dire les uns et les autres que l'expérimentation permet de faire des choses, de valider.

l'acceptation du report de six mois serait raisonnable et explicable aux interlocuteurs, qu'il s'agisse des opérateurs ou des collectivités locales. Sinon on ne comprendra pas qu'il faut tout faire en un an

Nous avons un certain nombre de points d'accord, au-delà des désaccords ponctuels sur tel ou tel amendement. Premier point d'accord : le dispositif Pinel est, comme tous les dispositifs fiscaux qui l'ont précédé, un dispositif de subventions par les dépenses fiscales- il coûte cher -, dont l'objectif est de construire dans les zones les plus tendues.

subissent des redressements fiscaux. Notre responsabilité consiste aussi à ne pas entraîner les contribuables vers des investissements mal orientés, peut-être du fait des mirages de la défiscalisation.

zone B2. Comme, dans les deux cas, l'établissement public de coopération intercommunale dispose de la compétence habitat, on est en droit de se demander si le priver de l'outil Pinel sera forcément la meilleure solution Surtout au regard des loyers de sortie dans ce type d'opérations, qui peuvent répondre aux besoins d'un certain nombre de familles. Je n'insiste pas sur la situation de ressources des habitants de ces futures métropoles. Le dispositif Pinel peut répondre à une demande assez précise de certaines familles : il convient donc de faire en sorte

Pour ma part, je me suis appuyé, avec la commission des finances, sur des échantillons de transactions. Nous avons retenu un taux de 15 %, qui s'appliquerait

dont il est question, cela importe du reste assez peu, vu qu'elle est exonérée d'office en cas de mutation. Nous avons donc juxtaposition de régimes divers, ce qui n'aide pas à la bonne compréhension du système. Nous proposons, pour ce qui concerne l'évolution de la valeur des biens objet de la cession, de retenir soit un système d'amortissement linéaire, soit un système progressif avec accélération relative du taux d'amortissement à la fin de la période de détention. Dans les deux cas, il s'agirait de revenir à la période de référence de trente Même schématique, la raison d'être de nos amendements est de renforcer la taxation des plus-values, alors que, dans les faits, nombre de logements aidés par certains dispositifs d'incitation à l'investissement locatif deviennent non taxables au titre des plus-values au terme des périodes d'engagement

tout programme de construction de logements intermédiaires doit comporter au minimum une surface de 25 % de logements sociaux, sauf dans les communes qui comportent déjà plus de 50 % de logements sociaux. Lors de l'examen du présent projet de loi de finances en première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui a pour objet d'abaisser de 50 % à 35 % le seuil d'exemption de cette condition. Or, comme cela a été rappelé tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat en première partie, une telle extension pourrait fragiliser le dispositif existant au regard du droit communautaire, lequel limite la possibilité pour les États membres d'appliquer un taux réduit de TVA aux opérations « de livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale Dans le contexte d'une remontée du taux de 5,5 % applicable au logement locatif social, le Gouvernement souhaite prendre le temps de s'assurer de la compatibilité de ces dispositions avec le droit communautaire et reporter leur entrée en vigueur au 1 janvier 2019. C'est pourquoi l'article

impôts, permet aux exploitants locaux de bénéficier de taux d'aide fiscale supérieurs aux dispositifs de réduction d'impôt et de déduction de base fiscale prévus aux articles 199 Les entreprises conservent aujourd'hui un droit d'option entre le dispositif du crédit d'impôt et le dispositif de la défiscalisation : dans tous les cas s'agissant du logement social ; dans le seul cas où leur chiffre d'affaires n'excède pas 20 millions d'euros s'agissant de l'investissement productif. Au-delà de 20 millions d'euros, les entreprises doivent obligatoirement opter pour le crédit d'impôt. La loi de finances initiale pour 2016 a prévu une extinction progressive de ces mécanismes l'abaissement du seuil de chiffre d'affaires à à 15 millions d'euros à compter du 1janvier 2018, à 10 millions d'euros à compter du 1janvier 2019 et à 5 millions d'euros au 1janvier 2020, à la condition que soit mis en place un

Il est donc indispensable, à l'instar de ce qui est aujourd'hui prévu pour les collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution pour lesquelles la date d'extinction des dispositifs d'aide fiscale est fixée au 31 décembre 2025, de prolonger les dispositifs applicables dans les départements d'outre-mer. il s'agit, d'une part, de donner de la stabilité et de la visibilité dans le temps aux investisseurs et aux exploitants sur des dispositifs essentiels au développement économique des outre-mer et, d'autre part, avant de le basculement de la défiscalisation vers le crédit d'impôt, d'engager une véritable évaluation de ces dispositifs. La parole

Nous envisageons de faire en sorte que les assises des outre-mer, qui se tiendront jusqu'au printemps 2018, soient l'occasion d'examiner les difficultés liées à ce préfinancement et d'étudier notamment le rôle des établissements de crédit il importe de trouver un accord pour garantir ledit préfinancement. Nous souhaitons aussi que les améliorations qui pourront être apportées au régime de défiscalisation mis en place pour soutenir les investissements en outre-mer soient ainsi confortées. S'agissant de la date de fin du dispositif pour les départements d'outre-mer, les régimes d'aide fiscale à l'investissement productif en outre-mer, qui constituent des aides d'État, sont aujourd'hui soumis à un encadrement européen et ne peuvent être prorogés en dehors de ce strict cadre. Ainsi, compte tenu de l'échéance des lignes directrices européennes afférentes aux aides à finalité régionale

Le législateur ayant fait le choix de systématiser le crédit d'impôt en remplacement de la défiscalisation, il convient de tirer les conséquences des premières expériences pour améliorer le fonctionnement de ce mode de financement, par ailleurs plutôt vertueux. En l'occurrence, on constate que ni Bpifrance ni les banques n'ont mis en place de dispositifs opérationnels de préfinancement, en particulier pour les petites entreprises. Elles ont donc recours au crédit-bail ou à la location longue durée avec option d'achat pour pallier leurs difficultés d'accès au crédit bancaire. C'est pourquoi le présent amendement vise à rassurer les prêteurs en mettant en place un mécanisme de cession de la créance de l'exploitant au prêteur. Il s'agit par ce biais d'apporter une garantie au prêteur en facilitant les formalités qui permettent à l'État de le rembourser directement. Quel

crédit-bailleresse risquerait d'entraîner une augmentation du coût de financement des investissements. Or il nous paraît nécessaire de préserver le crédit d'impôt de schémas qui seraient par ailleurs potentiellement abusifs. C'est donc davantage par souci de simplicité et de maîtrise des dispositifs que le Gouvernement est défavorable à l'amendement.

et que les enjeux de la reconstruction imposent la mise en oeuvre de dispositifs incitatifs afin de relancer l'activité, le présent amendement vise à faire bénéficier Saint-Martin d'un taux de réduction d'impôt majoré pour le bénéfice de l'aide fiscale à l'investissement productif, le même que celui qui est applicable aujourd'hui en Guyane et à Mayotte.

du dispositif de solidarité nationale au profit de la reconstruction de Saint-Martin. Quel est l'avis du Gouvernement ?

aux dispositifs d'exonération, pour tous les outre-mer les travaux qui répondraient à la remise en état d'investissements productifs en matière de logement social,

Afin de développer les énergies renouvelables, les investissements dans le photovoltaïque bénéficiaient avant 2011 de plusieurs dispositifs fiscaux : le crédit d'impôt développement durable, la réduction d'impôt sur le revenu dite « Dans les outre-mer, où le potentiel de développement de l'énergie solaire est considérable, ces investissements bénéficiaient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 et de la déduction d'assiette prévue à l'article 217 . Toutefois, en loi de finances pour 2011, au motif que ce mode de production d'électricité bénéficiait du système d'obligation d'achat à des prix avantageux, le législateur a décidé de restreindre les avantages fiscaux afférents pour éviter le cumul des aides publiques. En particulier, les investissements dans le photovoltaïque ont été exclus du champ de la défiscalisation outre-mer, du dispositif « Madelin et de l'ISF-PME. Paradoxalement, alors qu'il s'agissait d'éviter le cumul d'aides publiques, cette exclusion du champ des avantages fiscaux concernait également les investissements dans le photovoltaïque qui ne bénéficient pas des tarifs d'achat garantis, en cas d'autoconsommation, par exemple. Pour remédier à cette anomalie, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a rétabli les avantages fiscaux « Madelin » et ISF-PME pour les investissements dans le photovoltaïque qui ne bénéficient pas de tarifs d'achat garantis, en conformité avec le principe de non-cumul des aides fiscales pour une même activité. Elle n'a toutefois pas rétabli les avantages fiscaux spécifiques aux outre-mer. En cohérence avec la loi

se conformer au principe de non-cumul des aides publiques pour une même activité et rétablir l'égalité de traitement entre les différentes filières de production d'énergies renouvelables. Rappelons en outre que les outre-mer restent éminemment dépendants de l'importation d'énergies fossiles pour assurer leurs besoins au niveau énergétique.

Alors qu'elles disposent d'un immense potentiel d'énergie solaire, ces collectivités sont encore fortement dépendantes des énergies fossiles. Le dispositif que je vous propose permettrait de favoriser le développement des procédés de stockage de cette énergie,

sont les derniers comptes déposés à la date de mise en service de l'investissement, afin de réduire le risque de redressement fiscal pour les investisseurs. Quel est l'avis de la commission ? Notre collègue Michel

Pour bénéficier des avantages fiscaux attachés aux investissements outre-mer, il faut que l'entreprise qui effectue l'investissement et celle qui l'exploite respectent toutes les deux leurs obligations fiscales, sociales et commerciales. Cette mesure de moralisation et d'équité paraît légitime et il n'est pas envisageable de revenir sur ce principe. À la date de la réalisation de l'investissement, c'est-à-dire la date du fait générateur de l'avantage fiscal, il faut que l'entreprise chargée du financement et l'entreprise exploitante qui en bénéficie soient à jour de leurs obligations fiscales, sociales et commerciales. un texte fiscal n'a pas vocation à déroger à la législation commerciale. En particulier, les dates de dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce sont celles qui sont prévues par le code de commerce. Les sociétés concernées déposent leurs comptes auprès du greffe dans le mois qui suit l'approbation des comptes par l'assemblée, et ce conformément au droit commercial. Pour éviter toute ambiguïté et répondre à votre interpellation, la doctrine administrative pourra être précisée sur ce point. Je souhaite aussi préciser que la notion de « réalisation », qui figure dans votre amendement, permet de couvrir l'ensemble des faits générateurs concernés par le dispositif de défiscalisation et qu'il ne nous semble pas pertinent

prolonger le dispositif de réduction d'impôt en faveur de la construction de logements sociaux dans les départements d'outre-mer jusqu'en 2025, sociaux dans les départements d'outre-mer jusqu'en 2025, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution, en fixant au premier euro, afin de pouvoir totalement contrôler le dispositif et en limiter les éventuelles dérives.

Cet amendement, adopté dans un premier temps en commission des finances de l'Assemblée nationale mais non intégré au texte, vise à répondre aux besoins de réhabilitation, qui représentent sans aucun doute le principal enjeu de la période à venir. Pour ce qui est des opérations de réhabilitation, le crédit d'impôt n'est pas substituable à la réduction d'impôt, comme le montrent les différentes évaluations. Il s'avère que l'arrêt du dispositif de défiscalisation et le passage en crédit d'impôt empêcheraient la réalisation de nombreuses petites opérations de réhabilitation de logements sociaux, car des agences immobilières sociales n'ont pas droit au crédit d'impôt

cet amendement permet de ne pas mettre un terme à cette mesure, qui ne trouve pas d'équivalent au travers du crédit d'impôt. Elle permettra de poursuivre la lutte contre la vétusté du parc social, résultant en partie de conditions climatiques propres aux outre-mer. En outre, il y a lieu d'accélérer la mise aux normes des logements et la mise en sécurité des locataires. Enfin, le désamiantage du parc social représente aujourd'hui un enjeu d'intérêt général, du fait de l'exposition à un risque sanitaire majeur des populations. L'amendement tend, enfin, à élargir les travaux éligibles aux travaux de réhabilitation sismique ou paracyclonique. Ce dispositif viendrait s'inscrire en complément du crédit d'impôt, par ailleurs limité au secteur ANRU et pour lequel le montant des travaux est plafonné.

M. le rapporteur général

Cet amendement vise à maintenir constant le niveau d'aide fiscale accessible pour les projets d'investissement ultramarins éligibles à la défiscalisation à l'impôt sur les sociétés, dans le contexte de baisse du taux normal de cet impôt. L'aide fiscale à l'investissement outre-mer l'impôt sur les sociétés est un outil essentiel pour les porteurs de projets ultramarins, notamment dans la zone Pacifique, où le crédit d'impôt La trajectoire de baisse du taux d'impôt sur les sociétés pour toutes les entreprises à partir de 2019 aura un impact négatif certain sur le plan de financement des projets ultramarins qui prévoient d'avoir recours à la défiscalisation à l'impôt sur les sociétés, notamment les projets très structurants, dont le plan de financement doit souvent être bouclé plusieurs années avant la survenance du fait générateur de l'aide. Dans le même temps, les surcoûts subis par les porteurs de projets ultramarins, du fait de l'insularité et de la taille étroite de leur marché, restent inchangés, la défiscalisation ayant en principe pour objectif de compenser ces surcoûts. Il convient de rappeler par ailleurs que la baisse de l'impôt sur les sociétés ne profitera pas aux entreprises des collectivités d'outre-mer à autonomie fiscale, en particulier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour lesquelles les projets structurants sont, pour l'essentiel, financés par le dispositif prévu à l'article 217 du code général des impôts. Afin de ne pas handicaper lesdits projets structurants du fait d'une conséquence de la trajectoire de baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, l'amendement tend à inscrire le principe d'une base éligible inflatée du rapport entre le taux de l'impôt sur les sociétés en vigueur actuellement, soit 33,33 %, et les nouveaux taux normaux d'imposition s'appliquant pour toutes les entreprises à partir de 2019.

Cet amendement vise à maintenir constant le niveau d'aide fiscale accessible pour les projets d'investissement ultramarins éligibles à la défiscalisation à l'impôt sur les sociétés, dans le contexte de baisse du taux normal de cet

Le présent amendement a pour objet de favoriser le développement du secteur culturel dans les outre-mer. À cette fin, il vise, à compter du 1 janvier 2019, à assujettir systématiquement les entreprises, employeurs et organismes exerçant dans le domaine de la culture et du patrimoine au régime bonifié d'exonération de cotisations sociales. également à augmenter les réductions d'impôt dont peuvent bénéficier les particuliers ou les entreprises au titre du mécénat. Quel est l'avis de la

De fait, orphelins de l'ISF, les investisseurs les plus aisés se sont retrouvés à imaginer un nouveau dispositif d'accueil de leurs investissements au moins aussi rentable. L'ISF-PME, par sa quotité et le niveau élevé de réduction d'impôt, aurait pu constituer l'instrument de la quasi-disparition de l'ISF. Il n'en fut jamais rien. Il n'en fut jamais rien. Dans les faits, ce sont des versements au capital de sociétés non cotées, ou au bénéfice de fondations diverses, pour un montant de 1 milliard d'euros environ. Loin, donc des 900 milliards d'euros empruntés chaque année aux banques par les entreprises du secteur non financier et pour un coût plus élevé pour les finances publiques, chacun en conviendra. Les redevables de la première tranche ont déclaré un patrimoine imposable de 450 milliards d'euros et réalisé des investissements pour 450 millions d'euros, soit un taux d'« effort » de 0,1 %. L'ISF-PME a toujours tourné autour du milliard d'euros, bon an mal an, engendrant un faible effet de levier et une forte dépense fiscale, au regard des sommes ainsi collectées. L'objectif de l'article 39 est donc de renforcer le plus ancien dispositif, le dispositif Madelin, ce qui explique que certains amendements tendent à relever le seuil d'application maximal

ni le Madelin, pourtant beaucoup plus ancien, ne semblent vraiment avoir atteint leur objectif, si ce n'est du point de vue immédiat de la réduction d'impôt, et donc de la baisse des ressources pour le budget de la République. Quel

Le présent amendement vise donc à porter la réduction d'impôt à 30 %, ce qui nous paraît raisonnable, au lieu des 25 % proposés par l'Assemblée nationale, en la plaçant sous le plafonnement global de 18 000 euros contre les 10 000 euros actuels.

Créés par la loi du 1 août 2003 pour l'initiative économique, les fonds d'investissement de proximité, ou FIP, sont des véhicules qui doivent investir 70 % de leur actif

En 2007, le législateur, constatant qu'aucun des FIP levés depuis quatre ans n'avait choisi d'investir en Corse, a créé le FIP-Corse. Ce véhicule devait, grâce à un dispositif fiscal plus avantageux que sur le reste du territoire français- 50 % de déduction fiscale pour les FIP-Corse, contre 25 % pour les FIP continentaux -, orienter l'épargne des Français et mettre enfin la Corse sur la route de la finance. Dix ans se sont écoulés, et nous pouvons, à la lumière des chiffres, considérer que le dispositif a largement atteint ses objectifs. Les montants collectés une quinzaine de fonds, gérés par cinq sociétés de gestion différentes, se montent aujourd'hui à près de 380 millions d'euros. On estime que les sociétés financées par les FIP-Corse représentent 2 000 emplois directs en Corse et 7 000 emplois si on y ajoute les emplois induits. Les FIP-Corse ont parfaitement répondu à l'objectif fixé de mettre fin à l'exclusion de la Corse des activités de capital-investissement. Mais, faut-il le rappeler, cette intégration reste très fragile, car elle est le résultat d'un avantage fiscal qui incite l'épargnant à orienter une partie de son épargne vers la Corse. Aujourd'hui, les taux de réduction actuels sont de 38 % pour la souscription d'un FIP-Corse, contre 18 % pour un FIP finançant les entreprises continentales. Niveler cet avantage à tout le territoire français revient à refaire de la Corse un désert financier.

Pour rester attractif, le FIP-Corse doit nécessairement maintenir son différentiel de 20 points par rapport aux FIP nationaux. L'Assemblée nationale ayant porté pour 2018 le taux général de 18 % à 25

Il nous semble important de rappeler que les activités immobilières sont exclues du champ des activités que peuvent exercer les PME dont les parts sont éligibles à la réduction d'impôt « Madelin », et que, lorsqu'une PME a une activité commerciale, et non immobilière, elle est alors éligible à la réduction d'impôt « Madelin ». Cette distinction entre activité immobilière et activité commerciale constitue un principe fiscal présent dans de nombreux autres dispositifs et qu'il convient de préserver. En outre, au regard du bénéfice de la réduction d'impôt « Madelin », il ne serait pas justifié de traiter des activités de nature commerciale différemment des autres activités de même nature. Une telle différence de traitement, faute d'être suffisamment justifiée, serait susceptible de constituer une rupture d'égalité. Enfin, cette distinction paraît utile dans les discussions que nous avons avec la Commission européenne à propos du respect des exigences en matière d'aides d'État.

Merci